de l'article 1 reporte la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la mise en place de la juridiction unique des injonctions de payer. Un report est en effet la moindre des choses, mais, plus qu'un report, nous souhaitons un recul, car, selon nous, cette juridiction ne devrait tout simplement pas voir le jour. La création de cette juridiction va à l'encontre du projet de société que nous portons. Elle favorisera davantage encore les compagnies d'assurances ainsi que les banques, qui émettent

des sommes considérables et peuvent parfois ruiner des vies entières, le tout dans une logique purement gestionnaire. Rappelons que nous nous étions déjà opposés à cette

portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs. Cette entrée en vigueur, initialement prévue le 1 octobre 2020, est reportée au 31 mars 2021. Un texte de ratification de cette ordonnance aurait dû être présenté au Parlement l'été mais, en raison de la crise sanitaire que nous connaissons, le Gouvernement a repoussé l'échéance, dans un souci de faisabilité matérielle. Nous nous sommes déjà exprimés pour dire notre désaccord quant au fond, désaccord d'autant plus important qu'il s'agit d'une refonte du code pénal pour les mineurs par voie d'ordonnance. En réalité, ce que vous proposez, madame la garde des sceaux, c'est de faire davantage avec des moyens absolument indigents pour la justice des enfants, dans le cadre d'une accélération de la répression pénale,

protectrices pour tous, professionnels comme usagers, et se trouvent de fait fortement ralentis, voire à l'arrêt dans certains territoires, au détriment de l'accompagnement éducatif des enfants ». Pour toutes ces raisons, nous demandons, non un report, mais carrément l'abandon du texte.

dont la préparation va durer très longtemps- plus longtemps que l'élaboration d'un projet de loi -, et nous parler d'un vaste débat pour la ratification, alors que celle-ci n'est pas inscrite à l'ordre du jour, ni à l'Assemblée nationale

que ce serait une bonne chose si vous nous disiez ce soir que, par respect pour le Parlement, sur un sujet aussi fort, aussi sensible, on aura un débat parlementaire.

il importe que nous puissions mettre à niveau l'ensemble des stocks existants dans les tribunaux pour enfants. Pour cela, nous avons pris les moyens nécessaires : au 1 septembre

à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Vous le savez sans doute, lorsque nous rencontrons des représentants d'intérêts, il faut l'inscrire dans un répertoire numérique national.

Donnons-nous un petit peu de temps ; on peut penser que l'idée est juste- en vérité, les ayatollahs de la transparence nuisent parfois à la bonne économie locale -, mais commençons par bien tester l'affaire à l'échelon des parlementaires, à l'échelon national, avant de l'étendre aux collectivités territoriales. Donnons-nous deux ans

trop d'information nuise à l'information, puisqu'on ne pourra plus lire les informations intéressantes. Enfin, cette loi a été prévue pour qu'on puisse tracer l'impact du travail des lobbies sur l'élaboration de la norme. Autant il est normal que l'on suive le travail des parlementaires, des cabinets ministériels et de la haute administration, autant on peut s'interroger sur l'intérêt de tracer les rapports entre les représentants de terrain et les élus locaux pour l'élaboration de la norme, puisque ces derniers sont encadrés par celle-ci et ne participent pas du tout à son élaboration. Ils sont déjà encadrés par tout un ensemble de règles, notamment celles des marchés publics, pour évoquer les choses les plus sensibles, mais également toutes les lois qui traitent du fonctionnement des collectivités. C'est pourquoi il nous a paru raisonnable de proposer cet amendement, que je soutiens.

quand il n'y a pas le temps, quand les conditions ne sont pas réunies, il faut savoir se donner un délai pour que la loi soit bel et bien efficace et appliquée. Il ne faut pas dire « ce sera

des trois objectifs assignés à ces agences : la résorption du retard caractérisé d'équipements des quartiers et la lutte contre l'habitat indigne, la régularisation des habitations sans titre de propriété construites sur la zone des cinquante pas géométriques et le transfert de la gestion de la zone urbanisée de l'État aux collectivités locales. Sans cette concertation et sans mesures complémentaires, un report d'un an ne ferait, selon nos collègues, que repousser les problématiques liées à ces zones particulières. Si l'on prend le cas de la Martinique, il y a 7 000 constructions non encore régularisées et il reste à réaliser entre 250 millions et 300 millions d'euros de travaux d'équipement de base, tels que l'assainissement, l'accès à l'eau potable ou les routes d'accès aux quartiers de la zone des cinquante pas géométriques. Nous demandons, avec avec nos collègues, une action rapide de l'État sur ce sujet particulier.

présenter l'amendement n° 99 rectifié. L'envergure du plan de soutien à la filière automobile, présenté cette semaine par le Président de la République, répond à une réalité ; la filière automobile a été particulièrement ébranlée par la crise sanitaire, d'où ce plan de 8 milliards d'euros annoncé. Dans ce contexte, certaines adaptations paraissent nécessaires, et ce projet de loi s'y prête. Ainsi, en application de la loi du 5 mars 2007 et en conséquence d'un communiqué du CSA du 20 décembre 2018, la vente aux particuliers de véhicules équipés de la radio numérique terrestre devrait être obligatoire à compter du mois de juin prochain. Or le stock de véhicules n'intégrant pas ce dispositif technique et dont l'écoulement a été perturbé par la crise sanitaire reste très important. C'est pourquoi nous proposons de reporter de six mois l'application de cette obligation, afin de permettre la poursuite de la vente de modèles non équipés jusqu'au mois de décembre. La parole

pour présenter l'amendement n° 45 rectifié. La crise sanitaire affecte la mise en place du système de cotation rendu obligatoire dans les territoires visés par la loi ainsi que la mise en conformité des conventions de réservation qui ne portent pas exclusivement sur un flux annuel de logements. En effet, la mise en place de la cotation nécessite un travail transversal des acteurs participant à la réflexion sur les modalités de sa mise en oeuvre, définies dans le plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs : intercommunalités, communes, bailleurs sociaux. Dans les circonstances actuelles, ce travail de concertation est plus compliqué à initier. Pour ce qui concerne la mise en conformité des conventions de réservation, les bailleurs doivent tout d'abord informer simultanément tous les réservataires de la localisation, du nombre et des typologies de logements sociaux réservés par réservataire, dans le département. Il est ensuite nécessaire d'entamer une étape de négociation avec tous les réservataires, avant de signer de nouvelles conventions. Si celles-ci ne sont pas transmises avant la date du 24 novembre 2021, fixée par le décret du 20 février 2020 relatif à la gestion en flux des réservations de logements locatifs les logements réservés en stock s'ajoutent au flux annuel de logements réservés par l'État, jusqu'à la conclusion d'une convention conforme. Compte tenu du risque de sanction encouru par les bailleurs, qui n'auraient pas, en raison du contexte actuel de crise, finalisé leurs négociations, il semble plus raisonnable et plus efficient

parole est à M. le ministre. L'article 179 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite « loi ÉLAN », a rendu opposables, à partir du 1 janvier 2021, les diagnostics de performance énergétique. Il est proposé de prévoir l'entrée en vigueur de l'opposabilité des DPE au plus tard le 1 juillet 2021, soit un décalage d'une durée maximale de six mois. Cette date pourrait être avancée par décret si la situation le permettait. En effet, les filières professionnelles concernées, en particulier celle des diagnostiqueurs, devront à la fois assurer la reprise de l'activité des transactions immobilières dans les plus brefs délais, après un arrêt important de l'activité, avec la fragilisation qui en résulte, et se former aux nouvelles pratiques imposées par la réforme. Il nous semble que ce délai de six mois supplémentaire est nécessaire compte tenu de la difficulté créée par la situation sanitaire liée au Covid-19.

Sans publicité, la sincérité de ce tirage au sort n'est pas garantie. Le présent amendement vise à supprimer une disposition qui a pour effet de couvrir rétroactivement d'éventuelles nullités de procédure tirées de ce que la publicité de certains tirages au sort de jurés d'assises n'aurait pas été assurée. Une telle disposition ne peut se justifier. Les règles de procédure- celle-ci, en particulier -visent à garantir un procès équitable aux intéressés. Leur violation se fait donc nécessairement au détriment de la défense de l'accusé. On ne saurait justifier que cette dernière pâtisse du non-respect des règles de procédure par ceux qui sont chargés de procéder au tirage. En outre, cette disposition apparaît contraire au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Pour ces raisons, il convient de supprimer cette disposition. Quel

de sécuriser des procédures de tirage au sort des jurés, au moment où nous avons particulièrement besoin de pouvoir être certains que les sessions des cours d'assises se tiendront dans de bonnes conditions. C'est vraiment une question de sécurisation juridique liée au contexte particulier de crise. Il n'y a absolument aucune atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale.

concrètement dans ces juridictions considèrent qu'elles fonctionnent bien. L'audiencement devant la cour criminelle garantit un temps d'audience suffisant pour examiner les affaires comme elles le méritent, le méritent, les accusés déjà renvoyés devant les cours d'assises ne peuvent être jugés par une cour criminelle qu'avec leur accord et le taux d'appel des arrêts rendus par les cours criminelles départementales est moins élevé que celui des cours d'assises.

aux justiciables, victimes comme accusés, d'obtenir des réponses plus rapides et tout aussi pertinentes dans l'affaire dans laquelle ils sont parties prenantes. Troisièmement,

Je pense que le Parlement aurait une responsabilité particulière si nous ne mettions pas en oeuvre toutes les solutions permettant d'éviter un enlisement des cours d'assises et la correctionnalisation des affaires qui pourrait en résulter, au détriment des victimes. Comme l'avait justement souligné le rapporteur François-Noël Buffet lors de l'examen de la loi de programmation et de réforme pour la justice, « l'allongement préoccupant des délais de jugement aux assises nécessite de rechercher des solutions innovantes » et « l'encombrement des assises conduit à la correctionnalisation massive de certains crimes, en matière de viol par exemple, ce qui ne permet pas de sanctionner ces crimes au niveau qui convient ». Sur cette base, votre nous avait apporté son appui. Les cours criminelles constituent donc une réponse solide, bien que toujours expérimentale à ce stade. Je vous propose que cette solution innovante puisse être mise à profit

effet, vous n'avez pas pu ignorer les débats qui ont eu lieu notamment au sein de notre commission. Votre raisonnement pose de nombreux problèmes.

vous aviez depuis le début l'intention d'acclimater une nouvelle manière de procéder au jugement des criminels. Cette question

Elle repose sur des fondements solides. Nous n'avons pas l'intention de l'abandonner pour des motifs de convenance judiciaire.

très angoissants pour l'exercice de la justice. Pour autant, si nous entrons, à la faveur de la crise sanitaire, dans un processus d'accélération de l'élimination des cours d'assises, pour les remplacer

être relaxés, un jugement professionnel à un jugement en humanité. Je ne dis pas que les magistrats ne sont pas capables d'humanité. Dieu merci, ils le sont le choix du jury d'assises, c'est le choix de Français désignés parmi les Français, c'est le choix du citoyen-juge,

d'assises. Face aux difficultés qui vous assaillent pour juger les criminels en France, il ne faut pas perdre de vue ces principes essentiels, qu'aucun de nos prédécesseurs, dans le Parlement de la République, n'a jamais abandonnés.

de la justice, nous ne pouvons pas accepter cette évolution. Je veux dire à mon tour que le groupe communiste républicain citoyen et écologiste est opposé à cette mesure et à la méthode que le Gouvernement utilise pour l'imposer. Madame la garde des sceaux, avant d'envisager de modifier en profondeur la façon dont la justice doit être rendue dans ce pays, il faudrait d'abord dresser le bilan des neuf expérimentations qui ont été conduites. Selon nous, la justice doit être rendue par le peuple.

les difficultés que nous rencontrons. Nous n'avons pas du tout l'intention d'abandonner la justice des cours d'assises, fort au contraire. C'est une justice essentielle. C'est la justice du peuple français.

urgence. L'article 12 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 a prolongé de deux mois la durée de validité de certaines ordonnances de protection

une récupération plus rapide des pensions alimentaires pour les personnes qui en sont privées. Celui-ci devait entrer en vigueur le 1 juin. Or il est reporté aux calendes grecques. Je n'ai même pas vu de date. On nous explique que c'est à cause de la crise sanitaire que ce dispositif n'est pas prêt.

alimentaires qui devait être progressivement déployé à compter du 1 juin 2020. Le report ne concerne que la première phase de la mise en oeuvre,

seulement des familles sont concernées. En attendant, celles qui font face à un impayé de pensions peuvent toujours recourir à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions qui continue d'exercer ses missions. Pour apprécier l'opportunité du report, j'ai interrogé les services du ministère des solidarités et ceux de la CNAF. Les CAF ont bien recruté les personnels supplémentaires pour assurer le service d'intermédiation, mais une partie de

La mise en oeuvre du dispositif nécessite aussi des échanges d'informations entre les tribunaux et la CAF. Sur ce point, les travaux de développement informatique ont été suspendus

De plus, l'activité partielle n'aura pas d'impact sur le budget des activités sociales et culturelles des CSE. En effet, le code du travail prévoit que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales ne peut pas être inférieure aux dépenses sociales de la meilleure des trois dernières années.

l'État prendra ses responsabilités vis-à-vis des établissements concernés, c'est-à-dire accordera les financements nécessaires aux prolongations de contrat.

Il est absolument essentiel pour la recherche française et pour le rayonnement de nos universités de leur permettre de reprendre leur travail. Toutes et tous ont besoin de cette prolongation de contrat.

c'est un point fondamental -est que toutes les demandes soient traitées de manière homogène sur le territoire national. Il ne faut pas qu'il y ait des traitements spécifiques par université. Pour ce faire, la conférence des présidents d'université vous demande que les moyens financiers destinés à cette prolongation ne fassent pas prolongation ne fassent pas l'objet d'une négociation « de gré à gré » entre le ministère et chaque établissement ; elle souhaite que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche définisse une enveloppe budgétaire spécifique. Encore

il y a l'obligation d'un nombre minimum d'années de thèse. Vous ne pouvez vous présenter à des concours qu'à la condition d'avoir passé votre thèse en deux ans ou trois ans.

autour de 100 millions d'euros. Ce n'est pas une petite somme pour l'enseignement supérieur. Je vous rappelle que votre collègue ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, a promis que, dans un élan budgétaire historique, elle abonderait le budget de la recherche en 2021 d'une somme de 400 millions

Il doit également faciliter le travail de traitement des établissements en leur accordant plus de temps, dans une période où leurs effectifs sont déjà très largement mobilisés par la crise sanitaire actuelle, puis par la préparation de la prochaine rentrée. Avec votre permission, monsieur le L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet, notamment dans les relations entre l'administration et ses agents, ou si la demande présente un caractère financier, ce qui est le cas en l'occurrence, puisque tous les contrats concernés par cet article sont rémunérés. Comme la demande de prolongation doit être présentée à l'administration au plus tard le 10 juillet 2020, date à ce jour de la fin de la période d'état d'urgence sanitaire, nombre de décisions implicites de rejet pourraient survenir d'ici au 10 septembre 2020, alors que les universités seront fermées au mois d'août. Afin de permettre un traitement serein et équitable des demandes de prolongation d'un contrat doctoral ou d'un contrat de recherche, le présent amendement vise à ce que les établissements disposent d'un délai de trois mois pour répondre avant que leur silence ne puisse être considéré comme une décision de rejet. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements

est favorable aux doctorants contractuels et aux bénéficiaires d'un contrat de recherche comme aux instances dirigeantes des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, qui auraient un délai supplémentaire avant que l'absence de réponse à une demande de prolongation ne devienne une décision implicite de rejet. En conséquence, l'avis est favorable.

qu'ils puissent être exonérés du paiement des droits d'inscription pour l'année supplémentaire qui sera nécessaire à la préparation de leur doctorat. La parole est à M.

de l'OCDE dans lequel le nombre de docteurs baisse tous les ans depuis dix ans. C'est évidemment un signal catastrophique pour notre recherche. S'inscrire en thèse, c'est lourd financièrement, l'équivalent de 500 euros en

sur toute cette période, sans qu'il soit besoin d'y ajouter l'exonération de droits d'inscription pour la prochaine année universitaire. Par ailleurs, une telle exonération, réservée aux seuls doctorants contractuels prolongés, me semble discutable en termes d'égalité de traitement et d'égal accès à l'instruction, des principes encore rappelés

technique un peu complexe. Quand vous êtes en dernière année de thèse, vous avez l'obligation de soutenir votre thèse avant le mois de décembre. Si vous ne le faites pas,

à M. Joël Guerriau. Cet article dispense, pendant toute la période d'état d'urgence sanitaire, un opérateur économique de l'obligation de notifier à l'acheteur public son éventuel placement en redressement judiciaire. En temps normal, l'acheteur public peut suspendre l'exécution d'un contrat dès lors qu'il est informé que l'exécuteur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire sans en avoir notifié l'acheteur. Quel est l'avis de Quel est l'avis de la commission ?

il ne déroge ni à l'article L. 2195-4 du code de la commande publique ni aux dispositions du code de commerce. L'objectif de l'article 1 est uniquement de faire obstacle à la possibilité

en effet exclues de tout effacement dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, ce alors même qu'elles sont prises en compte dans d'autres procédures. Cela comporte plusieurs effets pernicieux à notre sens. Premièrement, les débiteurs concernés se trouvent incités à privilégier d'autres mesures de traitement du surendettement que cette procédure de rétablissement personnel. Deuxièmement, un privilège indu peut apparaître au profit des créanciers professionnels. L'exclusion des dettes professionnelles de la procédure de rétablissement personnel est d'autant plus problématique que cette procédure se caractérise par sa finalité de redressement. C'est pourquoi nous souhaitons, par le présent amendement, harmoniser la prise en compte des dettes professionnelles dans le traitement du surendettement des particuliers. Une telle mise en cohérence se justifie particulièrement dans le contexte que nous connaissons,

Laborde. L'amendement n° 98 risque d'apporter une mauvaise réponse à une vraie question, celle de la relance économique. Le présent sous-amendement vise donc à conserver les mesures de publicité, afin de permettre à toutes les entreprises de connaître les marchés en cours.

! Voire ministre ! Je ne dirai pas si souvent du bien d'un membre du Gouvernement, profitons-en

et afin de faire face aux conséquences économiques des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, cet amendement vise à accélérer et à simplifier des procédures du livre VI du code de commerce, qui traite des difficultés des entreprises. des entreprises. Peu de procédures collectives sont actuellement engagées, mais il pourrait en être différemment à brève échéance. De nombreuses défaillances d'entreprises sont, hélas ! à envisager. Notre droit des procédures collectives doit s'adapter, il doit être plus réactif et agile afin de permettre de sauver un maximum d'entreprises et d'emplois. Cet amendement tend à proposer à cet effet, jusqu'à la fin de l'année 2020, des dérogations temporaires et exceptionnelles à certaines dispositions fixées par le code de commerce relatives au redressement des entreprises. Dans une perspective d'accroissement significatif du nombre de faillites à venir, il s'agit de rendre les procédures collectives plus efficaces et plus rapides. L'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie poursuit le même objectif avec des dispositions applicables pour l'essentiel jusqu'à la fin de 2020. Cet amendement va, sur certains points, plus loin. Il propose, jusqu'au 31 décembre 2020- l'ensemble des délais prévus tant par l'ordonnance que par l'amendement auront sans doute vocation à être prorogés le moment venu -, d'accélérer un délai des plans de sauvegarde, de permettre à l'administrateur de se voir autoriser par le juge-commissaire, en cas d'urgence, à se fonder sur les déclarations du débiteur et les documents comptables existants et de permettre aux professionnels un accès simplifié et exhaustif aux données pour faciliter l'accélération des procédures collectives. Par ailleurs, il faut souligner que l'objectif de déstigmatiser les entreprises, dont l'activité s'est arrêtée du jour au lendemain de façon involontaire, non en raison d'une faute de gestion, mais de décisions de l'État, nécessite de permettre aux entreprises un rebond rapide. et plus rapides. L'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie poursuit ramène le délai au terme duquel est radiée du registre du commerce et des sociétés la mention d'une procédure collective, lorsque le plan arrêté est toujours en cours, de deux ans à un an. Cette disposition est certes d'ordre réglementaire, mais nous estimons qu'une réduction à six mois, voire trois mois, aurait été préférable afin de faciliter la reprise économique.

est à Mme Laure Darcos. À la suite des auditions menées pendant le confinement par la délégation aux entreprises du Sénat et afin de faire face aux conséquences économiques des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, la question de la reprise de tout ou partie des salariés d'un fonds de commerce qui serait cédé a été évoquée. amendement vise à assurer la préservation de l'emploi. Actuellement, il est juridiquement impossible au cessionnaire d'un fonds de commerce en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de reprendre tout ou partie des salariés de l'entreprise.

paradoxalement les mandataires judiciaires en quête de sécurité juridique à licencier tous les salariés avant de procéder à la cession du fonds de commerce en l'absence de plan de cession. Le système actuel favorise en réalité un « tout ou rien » en matière d'emplois qui risque d'avoir des effets désastreux à l'heure du déconfinement. Des milliers d'emplois sont en jeu, et ils pourraient être sauvegardés si la procédure était aménagée. Il convient donc de préciser l'article L. 642-19 du code de commerce afin de prévoir un maintien de tout ou partie des salariés de l'entreprise, malgré la cessation d'activité, en cas de cession du fonds de commerce.

et on peut la céder avec les contrats de travail, soit la liquidation a produit ses effets, et on ne peut alors céder que les actifs, c'est-à-dire les machines et les immeubles- dans ce cas, il n'est pas possible de céder l'entreprise, puisqu'elle n'existe plus et que les contrats de travail ont été résiliés. Je ne crois pas que nous devions revenir sur ce principe,

de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée, de fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD et de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable va à l'encontre des droits des salariés. Il en est de même concernant les contrats de mission. La possibilité de fixer, une convention d'entreprise, le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission, de fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats et de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable va à l'encontre des droits des salariés. Le dispositif pourrait être envisageable s'il se limitait à prolonger les relations de travail qui n'ont pu se dérouler dans les conditions attendues du fait de la suspension des contrats, notamment en raison du recours à l'activité partielle. le dispositif ne limite pas ces dérogations aux entreprises ayant eu recours à l'activité partielle. Cette possibilité d'ouverture de manière dérogatoire pour les contrats en cours de modification des dates d'échéance doit respecter le principe selon lequel un contrat court ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Cet assouplissement des règles va encourager la multiplication des contrats courts. Les plus précaires, déjà fragilisés par la crise sanitaire, vont être directement touchés par ces mesures. L'allongement des CDD ne doit pas devenir la norme, au détriment des CDI, qui sécurisent davantage les salariés.

En avril, 843 000 demandeurs d'emploi supplémentaires sont venus gonfler un taux de chômage déjà trop élevé. Par conséquent, il me semble que tout dispositif, même temporaire, est intéressant. C'est pourquoi je propose d'ouvrir la possibilité, sous réserve d'un accord avec les partenaires sociaux

de manière exceptionnelle et pour une durée limitée, déroger à certaines règles. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis favorable

ainsi libellé : La parole est à M. le ministre. Le Gouvernement est favorable au remplacement de l'habilitation qui figurait aux alinéas 27 à 29 de l'article 1 du projet de loi voté en première lecture à l'Assemblée nationale par des dispositions inscrivant directement dans la loi

Toutefois, cet article ne comporte pas une disposition importante et nouvelle- l'injonction administrative de restriction d'accès -et prive d'effet utile une autre disposition- la transaction administrative -, alors que ces dispositions avaient été adoptées en première lecture dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dit DDADUE.

Monsieur le ministre, vous m'avez tout à l'heure évité une inconstitutionnalité ; je voudrais vous en éviter une à mon tour. En effet, il me semble qu'il est de jurisprudence constitutionnelle constante que l'administration ne peut s'octroyer de tels droits et que la loi ne peut pas plus lui en octroyer. Pour ce type de sanction,

crise sanitaire. Une autre conséquence de cette crise a été le report du renouvellement des membres des conseils de prud'hommes et de la commission paritaire régionale interprofessionnelle. Il était donc indispensable de prendre des mesures d'adaptation. C'est ce qu'a fait la commission. Le présent amendement s'inscrit dans la même démarche, tout en proposant une modification de l'intervalle entre les deux prochains scrutins. L'objectif est d'éviter toute rigidité inopportune sur la date d'organisation du scrutin en fixant ce dernier au cours du deuxième semestre de 2024.

M. André Gattolin. Cet amendement vise à tirer les conséquences pour Mayotte du report prévu par l'ordonnance du 1 avril 2020 du renouvellement général des conseillers prud'homaux à une date fixée au plus tard au 31 décembre 2022. L'objectif est de prévoir plusieurs coordinations et adaptations afin de maintenir l'échéance de la création du conseil de prud'hommes de Mayotte au 1 janvier 2022, et non au 31 décembre 2022, cette installation étant essentielle et ayant déjà fait l'objet de trois reports. Quel

utiles aux armées qui seraient statutairement éligibles à l'avancement au cours de cette prolongation. Il s'agit de tenir compte de l'effet d'une promotion intervenue au cours de la prolongation de service au-delà de la limite d'âge sur la durée de service du militaire de carrière promu à un grade auquel serait attachée une nouvelle limite d'âge et de garantir un droit à la reconversion aux militaires de carrière réintégrés dans leur statut de militaire de carrière.

M. le ministre. Cet amendement a pour objet d'ajouter à la version rédigée par la commission deux éléments : l'intégration dans les services, ouvrant droit à pension, du temps de prolongation de service qui permet aux militaires d'achever les formations de reconversion suspendues par l'épidémie de Covid-19 et la garantie du maintien de l'intégralité du droit à la reconversion au militaire qui a accepté de cesser sa reconversion ou de la différer pour rester en service. Quel est l'avis de la commission

est à M. le ministre. La réserve civique permet l'engagement bénévole et occasionnel de citoyens étrangers résidant régulièrement sur le territoire français. Ses membres s'engagent dans des projets qui peuvent concerner différents domaines d'action : la solidarité, le vivre ensemble, l'éducation, l'insertion, la santé, le sport, l'environnement, la mémoire et la citoyenneté, la coopération internationale. Actuellement, ces missions sont bénévoles et ne peuvent concerner que des activités d'intérêt général au sein d'organismes publics. Compte tenu des circonstances exceptionnelles que nous connaissons, le Gouvernement souhaite que les missions relevant de la réserve civique puissent être exceptionnellement et temporairement proposées jusqu'à six mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire pour toute personne morale chargée d'une mission de service public. Elles pourraient être exceptionnellement élargies à des actions, notamment, de régulation de flux et de distribution de masques.

qui servent dans cette réserve civique puissent intervenir auprès des personnes morales qui exercent une mission de service public. La commission n'y est pas opposée, à trois conditions. Tout d'abord, il doit bien s'agir de missions de service public,

parole est à M. le ministre. Cet amendement reprend, en le complétant, le dispositif de l'ordonnance du 25 mars 2020 visant à prolonger l'indemnisation des demandeurs d'emploi qui arrivent à l'épuisement de leurs droits au cours de la période de crise sanitaire. Cet amendement inscrit en dur dans la loi des dispositions de cette ordonnance en procédant à plusieurs adaptations. Il a pour objet de différencier cette prolongation des droits en fonction du régime d'indemnisation dont relève le demandeur d'emploi et, ainsi, de tenir compte des difficultés spécifiquement éprouvées dans la période par les artistes et techniciens intermittents du spectacle pour reprendre une activité professionnelle. Pour ces intermittents du spectacle, l'amendement permettra, s'il est adopté, de garantir un maintien de l'indemnisation jusqu'au 31 août 2021, conformément aux engagements pris par le Président de la République. L'amendement reprend en outre la mesure de sécurisation juridique adoptée en commission tendant à sécuriser le maintien de l'indemnisation des demandeurs d'emploi dont les droits sont arrivés à échéance

devant sa télé. Grâce au virtuel, les membres de la commission de la culture ont pu se réunir aujourd'hui, se parler et se dire que c'était un amendement qu'il fallait soutenir.

Je tiens à le dire, monsieur le ministre, parce qu'il concrétise un engagement qui a été pris par le Président de la République. Vous le savez, tous les intermittents,

dans un esprit constructif. Je pense que le secteur culturel, les intermittents du spectacle et les habitants de Mayotte seront reconnaissants de ce travail de coconstruction qui fait honneur à la Nation.

vous nous aviez répondu, madame la ministre, que ce n'était pas le bon système et que c'était même peut-être impossible. Nous pensons le contraire : c'est un système qui peut fonctionner, qui va fonctionner, si nous l'accompagnons d'un schéma plus global. global. Nous avons déjà mis 415 milliards d'euros sur la table en prêts garantis par l'État, en chômage partiel- je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une nationalisation des salaires,

alors que, pendant trois mois, nous avons aidé nos entreprises, nous allons avoir des licenciements massifs. Nous proposons donc d'interdire les licenciements et d'accompagner cette interdiction de l'ensemble de ces dispositifs. Ensuite, il y aura un plan de relance économique. Nous avons déjà eu ce débat ici hier ou avant-hier, mais il faut le poursuivre. Il y a de vraies questions autour des prêts garantis par l'État.

Pour autant, quand on regarde autour de nous, depuis le début de cette terrible crise, on constate que des pays tout à fait raisonnables ont mis en oeuvre ces dispositions.

Il ne s'agit pas d'interdire tout licenciement dans toute situation, mais,, de réserver cette mesure aux entreprises du CAC 40, qui distribuent des milliards de dividendes, dès lors qu'elles reçoivent des aides de l'État.

une aide de 5 milliards d'euros au Gouvernement. Je ne sais si le chèque est déjà signé, mais, dans le même temps, la Régie annonce la fermeture d'un certain nombre de sites, notamment celui de Dieppe, dans lequel ont été investies des dizaines de millions d'euros dernièrement avec l'aide des collectivités territoriales. C'est un site qui compte 350 employés,

seraient en vigueur. On ne lutte pas contre les licenciements en proclamant une interdiction générale, mais en soutenant les entreprises en difficulté afin qu'elles soient en mesure de conserver leurs salariés. Or il peut arriver que ce soutien soit insuffisant et que les entreprises soient tout de même conduites à licencier certains salariés pour en conserver d'autres. De plus, je note que cet amendement vise tous les motifs de licenciement, y compris les licenciements pour motif personnel, par exemple pour faute. Je vois mal ce qui justifie cette interdiction absolue. Par ailleurs, je

n'a pas interdit les licenciements. Un décret prévoit seulement que les difficultés économiques liées au Covid-19 ne peuvent constituer à elles seules un motif de licenciement dans la mesure où un dispositif de chômage partiel existe. C'est différent.

Je note qu'une entreprise peut avoir fait des bénéfices une année, en avoir reversé une partie à ses actionnaires et se trouver aujourd'hui, en raison de la crise, contrainte de licencier pour ne pas disparaître, la crise étant particulièrement brutale. Les dividendes versés peuvent d'ailleurs être sans commune mesure avec les difficultés rencontrées du fait de l'épidémie. Cet amendement a une portée générale et ne semble donc pas pertinent. S'agissant des paradis fiscaux, le fait d'avoir des filiales à l'étranger n'a pas nécessairement d'impact sur la situation de l'entreprise en France. L'amendement n° à interdire que les licenciements économiques et uniquement dans les entreprises du CAC 40 ayant bénéficié d'aides de l'État. Je note qu'il introduit une rupture d'égalité injustifiée entre les salariés d'une entreprise du CAC 40 et ceux dont l'entreprise n'est n'est pas cotée ou est cotée sur une autre place boursière. Pour reprendre l'exemple cité par ses auteurs, cet amendement protégerait temporairement les salariés de Renault, mais pas ceux de Toyota. Il pose en outre un problème de sécurité juridique s'il doit s'appliquer rétroactivement depuis le début de l'état d'urgence Enfin, encore une fois, ce n'est pas parce qu'une entreprise a bénéficié d'une aide publique que sa situation est viable pour autant. Telles sont les raisons qui ont conduit la commission des affaires sociales à émettre un avis défavorable sur ces trois amendements.

bonne méthode législative. Pour autant, c'est le seul moyen que nous ayons trouvé pour vous alerter une nouvelle fois sur

Face à la crise actuelle, vous avez pris la décision de reporter au mois de septembre prochain la réforme de l'indemnisation du chômage, qui devait entrer en vigueur en avril. l'autre partie de cette réforme est déjà entrée en vigueur en novembre 2019, ce qui a déjà privé de leurs droits beaucoup d'allocataires. C'est pourquoi nous vous demandons,

Mme Monique Lubin. Combien d'entreprises n'ont pu faire aboutir une convention de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif depuis le début de l'état d'urgence sanitaire ? L'étude d'impact est muette sur le sujet. En quoi un assouplissement du cadre du prêt de main-d'oeuvre entre entreprises se justifie-t-il ? Aucun élément ne figure non plus dans l'étude d'impact

Le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif entre entreprises est un dispositif très spécifique, qui place le salarié dans une situation atypique : son contrat de travail n'est ni rompu ni suspendu, mais il doit travailler dans une autre entreprise, hors de son cadre habituel de travail. C'est pourquoi ce dispositif est très encadré par le code du travail. Ce que d'aucuns nomment « formalisme » garantit la protection des travailleurs. L'article 1 vise à « assouplir » le dispositif, c'est-à-dire à réduire la protection des salariés concernés.

En outre, l'avenant au contrat de travail ne fixerait plus les horaires de travail dans l'entreprise utilisatrice. Dès lors, rien ne garantit que le volume horaire hebdomadaire resterait le même pour le salarié prêté à l'entreprise utilisatrice.

le maintien de l'emploi et éviter le chômage partiel et les licenciements. Le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif est l'un des outils à la disposition des entreprises et des associations. Si elles sont confrontées à une baisse ou à une

cotisations sociales et frais professionnels -sont refacturés à l'entreprise utilisatrice pour garantir le caractère non lucratif : il ne s'agit pas d'organiser une sorte de nouveau marché du travail. malgré l'appui du ministère du travail et les conventions types mises à disposition, notamment les avenants aux contrats de travail disponibles en ligne, certaines initiatives se heurtent à des difficultés d'application du cadre légal dans un contexte d'urgence économique.

Nous avions présenté, mardi dernier, un amendement qui visait à permettre la mise en oeuvre d'un dispositif alternatif à l'activité partielle de manière à accompagner les entreprises durablement affectées par la situation sanitaire et économique.

Il nous paraît nécessaire de mettre très rapidement en place de nouveaux dispositifs de préservation de l'emploi et des compétences. Ces dispositifs permettront aux entreprises d'ajuster à la baisse leur capacité de production, en fonction de la demande, et de limiter les coûts économiques et sociaux, tout en préservant l'emploi et les compétences pendant cette période.

comporter des engagements en matière d'emploi en contrepartie des aides reçues ; il devra être homologué par l'autorité administrative, ce qui nous paraît tout à fait normal.

Il vise à apporter un accompagnement de plus long terme à des entreprises confrontées à une baisse d'activité durable, mais disposant de réelles perspectives de reprise. Dans ce cadre, l'indemnité d'activité partielle et l'aide versée par l'État et l'assurance chômage pourront être majorées

plus poussé en cas de plan d'activité unilatérale. Bien que le texte ne le précise pas, nous vous incitons à aller dans ce sens,

il fait reposer ce geste de solidarité sur les salariés, y compris les plus mal payés, alors que les titres-restaurant sont un avantage acquis lié au contrat de travail qui doit leur revenir.

remis au Parlement au plus tard au mois d'octobre prochain, et, d'autre part, les résultats de la concertation qui va être menée avec les acteurs économiques afin de définir au mieux les modifications qui doivent être apportées à cette ordonnance, notamment en ce qui concerne l'encadrement des promotions de volume. Dans la rédaction résultant du

Or le contenu précis des aménagements qu'il conviendra de prévoir pour ces dispositions ne pourra être défini qu'à la lumière de l'évaluation qui est en cours et fera l'objet du rapport précité et d'une concertation très approfondie avec l'ensemble des acteurs.

S'il est nécessaire de faire évoluer le cadre législatif actuel pour mettre en cohérence le droit et la pratique, l'extension des missions des VIA au domaine de la diplomatie d'influence prévue par cet article va beaucoup trop loin. La diplomatie d'influence mise en oeuvre par les chefs de poste et relayée par notre politique culturelle s'inscrit dans le temps long et demande de la continuité dans les actions menées. L'organisation d'un festival du film ou du livre francophone ou une programmation culturelle se préparent généralement un à deux ans avant la tenue de l'événement. Or la durée d'immersion des VIA est limitée : le renouvellement fréquent des effectifs est incompatible avec une telle mission.

disposition vise à donner une base juridique solide aux différents types de missions actuellement confiées aux VIA, en particulier dans les services informatiques et dans les services immobiliers, où la contribution de ces jeunes diplômés à des fonctions d'exécution sous l'autorité d'agents d'encadrement est très appréciée.

L'Association des vétérans des essais nucléaires, l'AVEN, souligne que, depuis la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, des critères plus stricts ont été instaurés, notamment en ce qui concerne la dose minimale de rayonnements ionisants reçus. Or l'article 2 du présent projet de loi prévoit d'appliquer les nouveaux critères pour l'instruction des demandes d'indemnisation faites auprès

et ceux qui sont provoqués par d'autres causes. C'est pourquoi au critère de « risque négligeable » a succédé celui du millisievert : il s'agit de l'unité

d'accélération et de simplification de l'action publique, dit ASAP, afin de préciser l'interprétation qui doit être faite de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Pour rappel, cette

ce vote. Faute, pour le législateur, d'avoir prévu expressément des dispositions transitoires pour l'application de cet article lors du vote de la loi, le Conseil d'État a jugé, dans deux décisions du 27 janvier, que ses dispositions n'étaient applicables qu'aux demandes présentées devant le Civen postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances. La situation qui résulte de ces décisions est caractérisée par une atteinte à l'égalité de traitement des demandeurs, ainsi qu'à la sécurité juridique de l'ensemble des décisions désormais prises par le Civen.

L'État ne détient pas leur trésorerie, il n'en prend pas possession, et les entités dont la trésorerie est centralisée peuvent l'utiliser à tout moment pour leurs dépenses. Si les collectivités territoriales se trouvaient spoliées par la centralisation de leur trésorerie, cela se saurait ! Je rappelle

Les régies d'avances et de recettes des collectivités territoriales déposent également leur trésorerie sur le compte du Trésor, puisqu'elles sont un service des collectivités locales, sauf lorsqu'elle est constituée d'espèces. Les offices d'HLM bénéficient d'une exemption, sur laquelle le Gouvernement n'entend pas revenir.

le Commissariat à l'énergie atomique. La critique formulée par la commission des finances du Sénat se concentre sur la portée très générale de l'habilitation. Il s'agit principalement de recenser les organismes qui devraient normalement entrer dans le champ du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et déposer leurs disponibilités sur le compte du Trésor. La mesure permettra donc de faire respecter ce principe tout en octroyant des dérogations. L'autorisation d'ouverture des comptes en dehors du Trésor est appréciée au regard de critères essentiellement opérationnels. Elle ne soulève aucune difficulté de principe ou de jugement en opportunité. La centralisation des trésoreries publiques produit des effets, mais il faut du temps pour s'y préparer,

remboursés. C'est une condition de la réussite du déconfinement. Monsieur le ministre, faites comme le Président de la République : enfourchez le tigre, et rendez les masques gratuits

qui vont se poser à la fin de la période de transition, quand le Royaume-Uni quittera l'Union européenne : l'une concerne la possibilité, pour un assureur britannique, d'honorer les contrats signés

Il s'agit donc d'autoriser le Gouvernement à prendre des mesures qui seraient éventuellement nécessaires, à la fin de cette période de transition, si aucun accord n'était conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

de l'étendue et de l'exhaustivité des mesures envisagées. En ce qui concerne les services financiers, une habilitation couvrant un domaine bien plus large avait été prévue

L'ordonnance du 6 février 2019, prise sur le fondement de cette loi, était explicitement destinée à parer à un tel scénario, qui ne s'est finalement pas produit. L'accord euro-britannique trouvé au titre de l'article 50 a rendu caduque cette ordonnance. Or les deux mesures envisagées par le présent projet de loi ne couvrent qu'une partie infime des questions qui vont se poser en matière de services financiers en cas de Brexit sans accord à la fin de 2020. Lors de sa récente audition par la commission des finances du Sénat, Robert Ophèle, le président de l'Autorité des marchés financiers, s'inquiétait précisément que le régime applicable à l'issue

attirer l'attention sur l'importance de la coopération en matière de défense que la France entretient de longue date avec le Royaume-Uni et de l'implication du Parlement, non seulement dans le suivi de cette coopération, mais également dans sa concrétisation.

mené à un approfondissement sans précédent de la coopération engagée en 1995 avec la déclaration de Christchurch, aussi bien dans le domaine nucléaire qu'en matière de projection de forces d'interopérabilité ou d'intégration industrielle. Cette coopération est aujourd'hui solide. Elle s'est développée dans un nombre important de secteurs qui font l'objet de nombreux contrats. Le dixième anniversaire des accords de Lancaster House doit être l'occasion d'un renouvellement des engagements, mais aussi d'une nouvelle réflexion sur la convergence stratégique, stratégique, l'achèvement du projet de force expéditionnaire conjointe et le développement des piliers de la coopération bilatérale dans de nouveaux domaines, comme la cyberdéfense, la stratégie spatiale, l'intelligence artificielle et la coopération dans la gestion des menaces hybrides. Réussir le sommet bilatéral prévu à cette date est d'autant plus nécessaire qu'avec le Brexit la France jouera un rôle pivot dans l'arrimage du Royaume-Uni à son ambition d'une défense européenne. Le Royaume-Uni reste également indispensable au maintien de son autonomie et de sa souveraineté stratégique. Dans cette perspective, il nous paraît essentiel que le Parlement, et en particulier le Sénat, puisse disposer de toute la latitude nécessaire pour exercer son rôle de contrôle vigilant de cette coopération et de son évolution. Le Gouvernement doit comprendre que le Parlement joue un rôle central dans le renouvellement de la confiance nécessaire à la poursuite de cette coopération. Il sait les liens étroits tissés par les commissions compétentes du Sénat avec leurs homologues britanniques et leur rôle dans le suivi des négociations du Brexit ces quatre dernières années.

a démontré, depuis le début de l'état d'urgence, sa capacité à légiférer dans des délais très brefs. Nous pensons que la négociation d'un accord international de partenariat est très éloignée du champ des dispositions à prendre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ensuite, la décision quant à la Ensuite, la décision quant à la durée effective de la période de transition sera prise le 1 juillet prochain. C'est à cette date que l'on pourra évaluer s'il est nécessaire ou pas de légiférer rapidement,

Comment voulez-vous légiférer sans connaître les mesures équivalentes qui seront prises par le Royaume-Uni ni le dispositif effectivement retenu au niveau européen ? Pourquoi donner une habilitation avant de connaître l'issue des négociations sur, par exemple, l'autorité de sécurité du tunnel sous la Manche ? En l'état actuel des négociations, rien n'est arrêté pour ce qui concerne les règles de concurrence équitable.

qui a, depuis quatre ans, exercé un contrôle permanent et vigilant sur le processus du Brexit et joué un rôle de pédagogie et de relais auprès de nos concitoyens, en particulier ceux concernés par les conséquences du futur accord. En conclusion, si nous avons déposé cet amendement de suppression, ce n'est pas pour empêcher le Gouvernement d'agir rapidement ; c'est parce que nous considérons que l'établissement de nouvelles relations avec le Royaume-Uni devra faire l'objet d'un projet de loi, qui permettra au Parlement de débattre et d'arrêter les dispositions nécessaires.

La France n'a privé aucun de ses parlementaires d'un quelconque droit d'information. Je tiens vraiment à l'affirmer, ayant l'impression que certains se sentent victimes d'un processus qui n'existe pas. Par ailleurs, il y a bien un lien entre le PEA, l'assurance-vie et les autres sujets de la négociation

si nous adoptions un délai de quinze mois, une partie des problèmes que vous rencontrez avec le délai de sept mois seraient susceptibles de se poser de la même façon. En effet, au bout de quinze mois,

Nous avons juste une différence d'appréciation avec vous sur la durée pendant laquelle nous vous laissons les mains libres pour prendre des ordonnances. Nous ne vous disons pas que, à l'expiration de ce délai

doit être conclu, vous aurez les moyens de prendre les mesures nécessaires par ordonnances et que, s'il ne doit pas être conclu, nous serons alors à votre disposition pour délibérer de nouveau et apprécier si, oui ou non, nous vous donnons la possibilité de conserver cette compétence législative pendant plus longtemps. Au fond, c'est ici notre seul point de débat. Nous sommes vraiment à vos côtés pour que les positions et les intérêts de la France et de tous les acteurs économiques que vous avez mentionnés soient défendus. Nous sommes tous unis dans cette négociation sur le Brexit, nous sommes tous sur le même bateau européen et nous avons tous intérêt

Par conséquent, vous n'avez pas à vous inquiéter. Le Sénat de la République est à vos côtés dans cette négociation, comme il est aux côtés de Michel Barnier, avec lequel nous sommes nombreux à avoir des contacts très étroits et amicaux.

traité sa demande d'habilitation à légiférer par ordonnances dans des délais extrêmement contraints. Nous l'avons fait pour que nous soyons prêts, collectivement, dans l'hypothèse d'un Brexit « dur » en mars. Nous sommes tout à fait capables de le faire de nouveau,

Certains pourront considérer que je suis « imprudent » de vouloir laisser la bride sur le cou au Gouvernement pendant une période aussi longue. D'autres me trouveront naïf,

mais j'ai la conviction que, au cours des prochains mois, nous en découvrirons d'autres. Par conséquent, ce n'est pas la fin de l'histoire

transition. Nous sommes tous convaincus, en effet, que ce tunnel est une infrastructure à la fois incontournable et symbolique ; elle voit passer plus de 22 millions de passagers par an et plus de 140 milliards d'euros de marchandises. Afin de préserver son bon fonctionnement, la priorité- je le dis ici très formellement -est bien de maintenir cette conférence intergouvernementale comme unique organe, binational, de gouvernance du tunnel. Nous n'envisageons donc la désignation d'une autorité nationale pour la sécurité ferroviaire de la seule partie française du tunnel que comme une option de repli,

dès lors que la mesure envisagée dans l'habilitation dépend de plusieurs conditions soumises chacune à des calendriers différents, qui ne peuvent être anticipés avec certitude. Il faudra réviser une directive européenne

puisque, pour l'heure, nous n'avons pas identifié les problèmes qui pourraient surgir et qui nécessiteraient, selon vous, de prendre des ordonnances.

Par correction envers les personnes qui ont écrit ce texte, je veux souligner que sa finalité est très claire : préserver la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité, des personnes morales établies au Royaume-Uni ou de droit britannique exerçant une activité en France à la date de la fin de la période de transition, ainsi que, sous la même réserve, des personnes morales établies en France, dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume-Uni. Le Conseil constitutionnel exige seulement, au regard de l'article 38 de la Constitution, que le Gouvernement indique la finalité et le domaine d'intervention des habilitations demandées, mais aucunement qu'il précise la teneur

la situation des ressortissants britanniques qui résident en France ou y exercent une activité selon les conditions que nous avons précisées.

de procéder aux éventuels ajustements nécessaires de manière exhaustive. Vous pouvez naturellement compter sur moi pour revenir aussi souvent que vous le jugerez nécessaire vous présenter les mesures qui auront été prises et vous informer de la manière dont elles auront été mises en oeuvre. Quel est Je crois que nous ne nous comprenons pas sur cet amendement, madame la secrétaire d'État. Il me semble que le délai pendant lequel le Gouvernement peut modifier son texte est purement et simplement le délai d'habilitation.

de vote. Compte tenu de la situation et en guise d'encouragement à trouver un compromis positif avec l'Assemblée nationale, le groupe La République En Marche votera ce texte. la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. La parole est à